le rapporteur. Cet article entend permettre aux organismes de protection sociale et aux administrations de l'État d'échanger les données nécessaires à la gestion des droits des bénéficiaires, notamment le versement des prestations pour lesquelles ils remplissent les conditions prévues par le code de la sécurité sociale et par le code de l'action sociale et des familles. Dès lors que le champ de l'article englobe certaines prestations, comme le adultes handicapés (AAH), qui ne sont pas financées par les régimes de sécurité sociale, cet amendement vise à supprimer la référence aux deux codes mentionnés afin d'intégrer toutes les prestations sociales dans cet échange de données.

parmi ceux pouvant fixer une pension alimentaire. Cet amendement de coordination rédactionnelle vise à inclure ce nouvel acte parmi ceux pour lesquels un décret en Conseil d'État fixe les conditions que doivent respecter la date de paiement et les modalités de revalorisation annuelle du montant de la pension versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales.

Il répète cependant des dispositions que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avait déjà prévues quant à l'information des femmes enceintes sur l'ensemble de leurs droits, dès lors qu'elles déclarent leur grossesse auprès d'un organisme de sécurité sociale.

monsieur le rapporteur, vise tous les organismes de sécurité sociale, pas seulement ceux qui sont débiteurs de prestations familiales, et plus particulièrement, dans son intention initiale, les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses de mutualité sociale agricole destinataires des déclarations de grossesse.

: La parole est à M. le rapporteur. Le présent article vise à inscrire dans la loi les modalités de versement et de détermination de la prestation d'accueil et de restauration scolaire versée par les CAF d'outre-mer et la caisse de sécurité sociale de Mayotte aux services de restauration. Ces modalités sont fixées chaque année par un arrêté interministériel, qui, en général, est publié tardivement. L'article permettra d'introduire plus de lisibilité dans le calcul et la revalorisation de cette prestation, en l'indexant sur l'inflation et donc d'introduire de la prévisibilité dans la dotation attribuée aux caisses pour financer cette prestation. Cet amendement tire les conséquences des objectifs du présent article, en supprimant la référence aux arrêtés interministériels annuels fixant le montant global des dotations.

sur l'article. Cet article est une réelle avancée pour la reconnaissance de l'exposition des travailleurs aux polluants, en particulier aux pesticides et aux produits phytosanitaires. Nous connaissons la difficulté, pour les personnes concernées, de faire établir un lien entre leur activité professionnelle et les maladies, notamment le cancer. Cette bataille est particulièrement complexe pour nos compatriotes ultramarins qui se battent depuis des années pour que soit reconnu le lien entre l'exposition au chlordécone et les cancers, notamment celui de la prostate, dont la prévalence est impressionnante aux Antilles.

en 1990 en France, mais par le jeu de dérogations, les Antillais y ont été exposés trois ans de plus, jusqu'en 1993- et à vrai dire, les populations le sont encore ! La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, Joël Labbé et l'ensemble des membres du groupe écologiste souhaitent rappeler l'avancée que constitue ce fonds d'indemnisation des victimes des pesticides, issu d'un travail parlementaire assidu mené notamment par Nicole Bonnefoy, en lien avec la société civile.

-, mais nous voulons interpeller le Gouvernement sur une question à laquelle les victimes attendent une réponse, à savoir la fiscalisation des indemnités reçues. Alors que les indemnisations des victimes salariées sont défiscalisées,

pour reconnaître la maladie professionnelle ne doivent pas être restrictives afin de ne pas laisser de côté un grand nombre de victimes. Enfin, nous souhaitons attirer l'attention sur l'indemnisation des riverains, malades à cause des pesticides. Les données scientifiques s'accumulent sur ces sujets et il nous faut avancer vite. Plus Plus globalement, c'est aussi la question de l'accompagnement de la sortie de l'usage de ces molécules qui est posée, quand on parle des victimes des pesticides. L'amendement

L'Anses s'est autosaisie en 2011 pour mener une expertise collective visant à identifier, évaluer et caractériser les expositions aux pesticides des personnes travaillant dans l'agriculture, afin de proposer des actions de réduction et de prévention. Par pesticides, il était entendu les produits phytopharmaceutiques ou biocides et certains produits de médecine vétérinaire, notamment antiparasitaires. Les conclusions de l'Anses ont été publiées en 2016. Elles montrent que le risque d'exposition des travailleurs agricoles aux médicaments vétérinaires utilisés en traitement antiparasitaire est avéré dans le cas des éleveurs ovins, lorsqu'ils ont recours à des médicaments destinés à être utilisés en bain, douche ou pulvérisation ou après utilisation lors de manipulations d'animaux ou de laine. Les molécules incriminées entraient dans la composition de médicaments vétérinaires anciens. De nouveaux médicaments vétérinaires antiparasitaires ont été développés depuis avec de nouvelles molécules et des formulations réduisant l'exposition du manipulateur. Ils ont obtenu une autorisation de mise sur le marché après que des études visant à les évaluer et à caractériser le risque pour les utilisateurs En conséquence, en dehors des spécialités vétérinaires antiparasitaires pour lesquelles l'Anses a établi le risque, il reste à définir quels autres antiparasitaires sont inclus dans la liste des pesticides qui, au sens du présent article,

dans le cadre de la procédure normale de reconnaissance des maladies professionnelles les tableaux 58 et 59 de maladies professionnelles du régime agricole. La première recouvre les produits phytopharmaceutiques et biocides, la seconde y ajoute les médicaments vétérinaires antiparasitaires. Les personnes qui se trouveraient exposées à ces médicaments ne bénéficient alors pas de l'harmonisation de l'instruction permise par le FIVP et, pour les exploitants, de l'amélioration de l'indemnisation, puisque son périmètre exclut les antiparasitaires. La détermination par décret, comme tend à le prévoir cet amendement, d'une liste d'antiparasitaires dangereux conduira nécessairement à réajuster celle-ci en permanence. Il s'ensuivrait un affaiblissement des garanties des assurés, qui ne bénéficieraient d'une reconnaissance de leur maladie professionnelle que dans des conditions difficiles. Si l'exposition à ces médicaments est d'une dangerosité variable selon les usages, il est du ressort des employeurs et des vendeurs de procéder aux explications nécessaires. Et quand bien même l'usage serait entouré de toutes les précautions nécessaires, l'exposition à des médicaments antiparasitaires dangereux serait toujours possible. La MSA mène déjà un travail de prévention important pour prévenir les risques. Demander aux agriculteurs de faire la preuve d'un usage conforme aux règles d'utilisation nécessiterait, outre que cela irait contre la présomption d'imputabilité qui caractérise la reconnaissance des maladies professionnelles depuis la loi de 1898, de mener un contrôle sur les agriculteurs- or, il serait inutile, s'il n'était pas massif. L'avis de la commission est donc défavorable.

La mesure est d'autant plus nécessaire à la lumière des reconnaissances de maladies professionnelles qui devraient intervenir en raison de l'exposition au chlordécone. La commission a donc émis un avis favorable

à l'instant Mme la rapporteure : les personnes non salariées des professions agricoles exerçant leur activité en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte relèvent des règles du régime agricole au même titre que les non-salariés des professions agricoles de métropole, des tableaux de maladies professionnelles du régime agricole, dont ceux relatifs aux pathologies liées aux pesticides prévues par les tableaux 58

le Gouvernement méconnaît la vie des travailleurs et force l'instauration de la protection sociale comme objet du dialogue social, alors même que l'ordonnance dont on va débattre lundi et qui régit cette négociation n'a pas fini son chemin réglementaire. Il faut donc absolument

pouvant être négociées par les plateformes avec leurs travailleurs constituent un cavalier social au sens de la loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale. Elles doivent donc être supprimées ; ce sera l'objet de l'amendement n° 227 de la commission que nous examinerons

accessoire. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a déjà prévu une possibilité d'affiliation au régime général en tant qu'assimilé salarié pour les particuliers exerçant des activités de prestations de services, d'achats et de ventes, dont les recettes sont sont inférieures à 1 500 euros par an, dans le but de limiter autant que possible les situations de polyaffiliation qui génèrent de la complexité et d'éviter à ces personnes la charge de la création d'une entreprise. Dans le cas des travailleurs des plateformes, l'option pour le régime général ciblerait essentiellement les personnes exerçant une activité indépendante les plateformes en parallèle d'une activité principale salariée- pourraient ainsi accumuler des droits dans un seul régime au lieu de deux. Ceux dont l'activité principale est exercée sous le statut d'indépendant resteraient bien sûr libres de rattacher les revenus de leur activité ponctuelle à leur activité principale auprès de la sécurité sociale des indépendants. La mesure proposée paraît donc à la fois adaptée à la diversité des situations des personnes concernées et à l'enjeu de simplification de leur protection sociale. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

les cotisations versées par les travailleurs pour le financement de leur protection sociale complémentaire soient exclues de l'assiette de la CSG et des cotisations sociales, afin de ne pas augmenter le niveau de leurs prélèvements

Monsieur le secrétaire d'État, il faut nous expliquer comment on peut organiser le dialogue social entre des gens qui, en théorie, n'ont aucune relation contractuelle.

à Mme le rapporteur. Une mission sur la protection sociale des travailleurs de plateformes, portant notamment sur leur couverture au titre des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP), a récemment été confiée à M. Jean-Louis Rey, inspecteur général des affaires sociales. Son rapport est attendu très prochainement. L'article 50 a pour objet de demander au Gouvernement de remettre au Parlement, au plus tard le 31 janvier 2022, un rapport sur l'amélioration de la couverture sociale contre le risque AT-MP des travailleurs de plateformes.

La remise d'un rapport au Parlement sur ces questions permettra de mettre en exergue les différents scénarios d'évolution de la couverture des travailleurs de plateformes contre le risque AT-MP.

pourra utilement éclairer la représentation nationale.

Dans les critères pour bénéficier de cette mesure, le Gouvernement a exclu de fait les artistes-auteurs, dont les revenus artistiques présentent un caractère accessoire par rapport à leurs revenus principaux. Ainsi, parmi les 220 000 artistes-auteurs, seulement 10 % rempliront les trois conditions cumulatives à savoir : ne pas avoir déjà validé quatre trimestres une activité principale distincte de l'activité artistique ; avoir gagné moins de 600 heures SMIC en 2020 ou en 2021 son son activité artistique ; avoir en moyenne, sur 2017, 2018 et 2019, un nombre de trimestres validé supérieur à celui de 2020 ou 2021. Nous espérons que le Gouvernement va accepter de revoir sa copie

Toute personne qui a exercé une activité salariée ou assimilée hors du territoire français depuis le 1 juillet 1930 peut racheter des cotisations. Pour ce faire, l'assuré doit avoir adhéré à l'assurance vieillesse volontaire ou avoir été à la charge d'un régime obligatoire français d'assurance maladie pendant une durée qui est aujourd'hui établie à cinq ans. Le présent amendement vise à étendre la possibilité de rachat des cotisations aux personnes ayant été affiliées à la Caisse des Français de l'étranger (CFE).

Cette souplesse permettrait aux personnes qui n'ont pas suffisamment cotisé, en raison de périodes de travail à l'étranger, d'améliorer le montant de leur retraite en acquérant des points supplémentaires au titre de certaines périodes de leur carrière. Quel

du coût du versement par les artistes-auteurs de leurs cotisations prescrites d'assurance vieillesse concerne uniquement les assurés connaissant des difficultés économiques. Le but est de mieux cibler les artistes

Il ne nous paraît pas pertinent de restreindre ainsi l'aide au rachat de trimestres, tous les artistes-auteurs, quels qu'aient été leurs revenus, ayant pu subir le défaut d'appel de la cotisation vieillesse plafonnée. Il convient aujourd'hui, dans des conditions fixées par décret, de tous les rendre éligibles à cette aide, afin que toutes les personnes concernées puissent au plus vite atteindre et sécuriser le juste montant de leur pension. J'ajoute que cette notion-

Nous ne partageons pas cette analyse. Ces caisses connaissent déjà les personnes en difficulté au titre de leur action sociale. Par ailleurs, si vous élargissez le dispositif pour prendre en charge un certain nombre de cotisations qui n'ont pas été perçues, comment allez-vous le financer ?

Cet amendement s'inscrit dans le cadre de la réforme de l'invalidité, qui était prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, et qui va prochainement entrer en vigueur. Celle-ci permettra de garantir aux pensionnés d'invalidité un gain en cas d'exercice d'une activité professionnelle : ils pourront en effet conserver l'intégralité de leurs revenus jusqu'au salaire précédant le

soumis à une règle spécifique qui ne leur permet de conserver qu'au maximum 50 % de leur pension d'invalidité. Avec cet amendement, ils pourront en conserver l'intégralité jusqu'à ce que leurs ressources atteignent le salaire précédant le passage en invalidité.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), qui contribue à réduire la pauvreté, fait l'objet de trop d'erreurs, de fraudes et connaît un taux élevé de non-recours.

Je rappelle à ce propos que le Sénat examinera, le 9 décembre prochain, la proposition de loi visant à assurer la revalorisation des pensions de retraite agricoles les plus faibles, qui prévoit notamment de renforcer l'information des assurés sociaux sur les conditions d'attribution de l'ASPA, ainsi que sur les procédures de récupération sur succession.

Les demandes devront ainsi être justifiées au premier euro devant le Parlement. Il s'agit d'un principe de base de bonne gestion des finances publiques, dont l'application de longue date pour les finances de l'État n'empêche le bon fonctionnement d'aucun opérateur.

Par ailleurs, nous proposons d'octroyer formellement à ces fonds et organismes les montants des dotations pour 2022 que le Gouvernement compte leur accorder, selon les informations transmises à Mme la rapporteure générale après la réunion d'examen de ce PLFSS par la commission

Le Sénat a clairement manifesté lors de leur discussion son intention de renforcer le contrôle du Parlement sur les dépenses de la sécurité sociale, en particulier sur celles qui devraient, par nature, être limitatives. Les dotations aux fonds et agences visées dans cet amendement en constituent l'exemple parfait. Plusieurs de ces structures étaient d'ailleurs financées par l'État sous le régime des crédits limitatifs avant d'être transférées à la sécurité sociale, souvent contre l'avis du Sénat.

d'opérateurs partiellement financés dans le cadre du sixième sous-objectif de l'Ondam. Actuellement, le montant de ces dotations est fixé par arrêté ministériel, pris à l'issue d'un dialogue de gestion entre le ministère de la santé et chacun de ces opérateurs.

l'évolution de la situation sanitaire nécessitait de relever en urgence la dotation de Santé publique France ? Faudrait-il revenir devant le Parlement ? Oui ! Vous comprenez bien que ce n'est pas possible

tout simplement parce qu'il n'était pas obligé de le faire, à l'inverse des lois de finances. Nous entendons donc, par ces amendements, apporter une réponse à cet état de fait particulièrement anormal dans une démocratie parlementaire. Les crédits des fonds et des agences, qu'ils soient financés par l'État ou par la sécurité sociale,

Quel contraste entre l'annexe 8 du PLFSS, qui donne pour ces structures des informations partielles sur les exercices passés, et la justification au premier euro des projets annuels de performance annexés aux lois de finances !

en matière d'investissement et de modernisation, conformément aux décisions prises dans le cadre du plan Ma santé 2022. Cet amendement vise à préciser que les établissements de santé élaborant et mettant en oeuvre une politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins, ainsi qu'une gestion des risques visant à prévenir et traiter les événements indésirables liés à leurs activités, peuvent recourir à ce fonds afin d'améliorer l'organisation et l'efficience des soins. Quel est l'avis de la commission ?

-commande de prendre des mesures de court et moyen termes. Il s'agit de promouvoir la possibilité, dans les centres et maisons de santé, de recevoir et soigner des patients pour de petites urgences. La télémédecine permettrait également d'effectuer un premier bilan avant un passage aux urgences, grâce à la réalisation de prises de sang et de radios en lien, si besoin est, avec les hôpitaux concernés. Or cette possibilité nécessite, prioritairement dans les territoires moins denses en médecine de ville et en structures hospitalières ouvertes jour et nuit, des investissements qui pourraient directement être profitables à tous. Cet amendement vise également à réaffirmer les vertus d'une médecine de proximité, dans laquelle les urgences peu lourdes peuvent être traitées de façon moins traumatisante et moins coûteuse pour la collectivité.

Nous connaissons tous l'attachement de notre ancien rapporteur général à la lutte contre les actes médicaux inutiles et redondants. La documentation sur ce sujet est déjà dense, dont un

ainsi à mettre en cohérence les prévisions de dépenses de la branche avec les rectifications introduites aux articles 19 et 20 pour les tableaux d'équilibre. Quel est l'avis de

pris connaissance de cet amendement tout à l'heure. Nous ne courons pas, dans cet hémicycle, après les dépenses nouvelles au regard du déficit déjà considérable de l'assurance maladie.

et malgré la petite rallonge de 0,5 milliard d'euros annoncée lundi par Olivier Dussopt, c'est bien 2 milliards d'euros en moins qui sont prévus pour 2022 par rapport à 2021.

Pour 2022, l'Ondam aurait donc dû être proposé plutôt autour de 250 milliards d'euros. Ce sont donc près de 14 milliards d'euros de ressources supplémentaires qui vont manquer cette année pour atteindre cette évolution dite « naturelle » des dépenses. Ce n'est pas exceptionnel : on déplore les mêmes chiffres depuis des années. L'Ondam prévu à l'article 56 est donc largement insuffisant par rapport aux besoins des établissements de santé et de la médecine de ville face aux retards accumulés depuis des décennies, puisque c'est toujours la même politique qui est mise en oeuvre. Pour l'ensemble de ces raisons, nous voterons donc contre cet article et contre l'amendement n° 1073 du Gouvernement, qui se contente de relever de façon insuffisante le niveau du sous-objectif « Dépenses qui a besoin d'être revalorisé. Nous ne souhaitons donc pas entrer dans une logique de redéploiement entre les différents sous-objectifs, car chacun d'entre eux est important. C'est pourquoi nous nous abstiendrons sur les amendements de nos collègues, même si nous souhaitons comme

ne prend pas en compte les surcoûts liés à la covid-19, mais intègre bien les conséquences financières du Ségur de la santé. Cette progression traduit donc l'engagement de ce gouvernement en soutien au système de santé, contrairement à

profession de catégorie A, sont rémunérés sur la base d'une grille salariale datant de 1991. En 2017, leur salaire net mensuel médian, un an et demi après l'obtention du diplôme, s'élevait à 1 680 euros. Alors que l'on ne cesse de reconnaître l'importance du soin psychologique, les rémunérations des psychologues restent faibles, malgré leur qualification à « bac plus 5 quelquefois complétée par un doctorat. Malgré les demandes réitérées de la profession, le Gouvernement maintient son refus de revaloriser les carrières des psychologues hospitaliers, au motif que ceux-ci ne disposent pas d'un statut de professionnel de santé dans le code de la santé publique. S'il nous faut préserver le statut particulier des psychologues, nous ne pouvons pas, face au besoin d'accompagnement psychologique, accepter la paupérisation de cette profession souffrant déjà d'un comme dans les établissements publics de santé. Notre amendement vise par conséquent à permettre la revalorisation des 16 000 psychologues de la fonction publique hospitalière, pour mettre fin à leur exclusion des revalorisations du Ségur de la santé.

les établissements publics de santé sont confrontés à une hémorragie de cette profession et qu'il faut, dans le contexte de la présente crise de la santé mentale, y remédier au plus vite. Les

maladie « considère qu'il existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'Ondam avec une ampleur supérieure à un seuil fixé par décret qui ne peut excéder 1 %, il le notifie au Parlement, au Gouvernement et aux caisses nationales d'assurance maladie. Celles-ci proposent des mesures de redressement

en lien avec la crise sanitaire. Ensuite, je rappelle l'engagement du Gouvernement d'accompagner les établissements de santé de manière pérenne, avec plus de 15 milliards d'euros de soutien à l'investissement et 7 milliards d'euros de revalorisation des salaires programmés dans le Ségur de la santé, mais aussi de manière conjoncturelle, pour leur garantir les moyens de fonctionner pendant la crise actuelle. C'est d'ailleurs l'objet des deux amendements de revalorisation de l'Ondam que je porte pour 2021 et 2022. Rappelons enfin que les moyens des établissements de santé sont déjà préservés par le protocole pluriannuel signé avec les fédérations hospitalières, qui continue de s'appliquer en 2022, sachant qui plus est que, pour la première année, aucune économie n'est demandée en construction à l'hôpital. Je mets aux voix l'amendement n°

Un cadre pluriannuel existe déjà pour les ressources des établissements de santé. Il serait donc opportun de tenir compte de cette possibilité pour l'ensemble de l'Ondam, sans attendre les conclusions des travaux en cours. L'amendement Mme Raymonde Poncet Monge. Les financements dédiés à l'investissement ont servi, depuis de nombreuses années, de variable d'ajustement à la régulation comptable des enveloppes insuffisantes après année. Ils ont ainsi évolué moins vite que celui-ci, voire ont diminué. Selon la Drees, ces investissements représentaient 3,7 milliards d'euros en 2018, après une baisse constante durant toute la décennie.

Le Gouvernement, semblant enfin entendre les alertes du secteur, a accru l'effort d'investissement pour 2022. Cela ne suffira pas pour autant à combler le déficit cumulé des investissements et ne garantit pas aux hôpitaux une enveloppe pérenne,

Par ailleurs, là où le Gouvernement avait retenu l'an dernier une dispense totale, je constate cette année qu'il a retenu la rédaction proposée par le Sénat dans le PLFSS 2021, à savoir une absence de mesures de redressement si, et seulement si le dépassement est directement imputable à la crise sanitaire. J'invite donc notre collègue Bernard Jomier à retirer son amendement et à se rallier à l'amendement n° 233 de la commission, qui, plutôt que de supprimer l'article, le complète avec une information renforcée des commissions des affaires sociales.

Lorsque le comité considère qu'il existe un risque sérieux que les dépenses d'assurance maladie dépassent l'objectif avec une ampleur supérieure à un seuil fixé à 0,5 %, il le notifie au Parlement, ainsi qu'au Gouvernement et aux caisses

Il indique que ces conventions doivent expliciter les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens de fonctionnement dont les branches et les organismes disposent pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à ces fins par chacun des signataires. Cet amendement vise à compléter les dispositions relatives aux modalités de gestion, en indiquant qu'en cas de déficit les organismes visés doivent préciser les conditions de retour à l'équilibre.

nous le demandons depuis le début de la discussion de ce PLFSS, avec un horizon à 15 milliards d'euros de déficit pour la branche maladie et tout autant de questions, René-Paul Savary l'a souligné, sur la branche vieillesse. Il serait préférable que la discussion ait lieu au Parlement, dans le cadre du PLFSS, plutôt qu'au détour de la signature des COG ! Surtout, c'est penser que les caisses ont un réel pouvoir de pilotage et de redressement autonome de leurs comptes,

Comme tous les ans, le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévoit un transfert de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) à la branche maladie au titre de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, en se fondant sur le rapport qui évalue, tous les trois ans, le coût pour la branche maladie de cette sous-déclaration. L'article 57 tend à accroître de 100 millions

L'augmentation de ce versement à l'assurance maladie, alors que de nombreux efforts ont été réalisés en matière de sous-déclaration, s'apparente de plus en plus à un détournement des excédents cumulés de la branche AT-MP au profit du rééquilibrage de la branche maladie. Si pendant les sept dernières années, au cours desquelles le transfert a été fixé à 1 milliard d'euros, on avait pris pour référence de ce versement la fourchette basse des estimations de la commission d'évaluation, soit en moyenne près de 800 millions d'euros, il s'en serait suivi un gain moyen pour la branche d'un peu plus de 200 millions d'euros.

depuis plusieurs années par la branche AT-MP et d'appeler à une augmentation des dépenses de prévention. En effet, les 100 millions d'euros restants pourraient judicieusement être utilisés pour financer des actions en ce sens, actions plus que jamais nécessaires dans le cadre de la prochaine convention d'objectifs et de gestion période 2023 à 2027. À moyen terme, il importe pour rééquilibrer la situation de la branche de diminuer les cotisations versées par les entreprises et, en gage, d'exiger d'elles

ne sortent pas de nulle part. Ils sont le fruit de travaux et d'évaluations. La commission chargée d'évaluer le coût de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles s'est réunie au premier semestre 2021.

augmentation de 100 millions d'euros par rapport aux transferts opérés depuis 2015 par la branche AT-MP, apparaît comme cohérent avec la trajectoire d'augmentation définie par le rapport de la commission, dont vous avez pris connaissance.

Nous souhaitons faire évaluer, par la commission instituée à l'article L. 176-2 du code de la sécurité sociale, le coût des pathologies psychiques liées au travail actuellement supporté par l'assurance maladie.

Comme le reconnaît elle-même la commission, les fragilités méthodologiques d'une telle évaluation, liées au caractère plurifactoriel de ces pathologies, sont inévitables. Sincèrement, il vaut mieux que les médecins du travail

qui ont tenu la ligne pour que notre pays résiste ? J'ai l'exemple d'une infirmière atteinte du covid-19 qui, son mari étant pneumologue, a fait le choix d'être soignée à domicile pour ne pas encombrer l'hôpital où ils travaillent tous les deux.

et le sentiment de ne pas être reconnus, sans compter qu'ils ont perdu, en plus de leur santé, une partie des primes annuelles auxquelles ils ont droit.

pour 1999, qui concerne le dispositif de retraite anticipée des travailleurs de l'amiante, et une éventuelle réparation des malades de la covid-19.

L'amiante n'est peut-être plus à la mode, mais elle est toujours bien présente dans nos murs et responsable, chaque année, de nombreux cancers.

et nous devrions donc, aussi, trouver une audience sur la partie gauche de notre hémicycle. Alors que cette réforme de 2014 porte la durée d'assurance nécessaire pour l'obtention d'une pension à taux plein à 43 annuités à compter de la génération 1973,

vous avez vous-même employé, ni d'ailleurs de façon uniforme, afin de prendre en compte les spécificités des parcours de vie et des aspirations de chacun, dans un esprit de renforcement de la liberté de choix. Par exemple, celui qui souhaite

des enjeux de simplicité, de lisibilité, d'équité entre assurés à travers le rapprochement de règles distinctes selon les différents régimes, en particulier entre les secteurs public et privé. Il convient aussi qu'une vie de travail offre une pension digne : toute retraite pour une carrière complète devra ainsi être supérieure à 1 000 euros par mois.

Au-delà du fond, sur lequel nous avons et nous aurons probablement quelques divergences, nous avons donc aussi une divergence sur le moment. Une telle réforme ne peut en effet être engagée qu'une fois la situation sanitaire totalement sous contrôle. être soumise à un intense débat démocratique, et je crois que celui-ci s'annonce. Quant à votre proposition de réunir de nouveau une conférence de financement-

que ce soit les vôtres, monsieur le rapporteur, ou celles du Gouvernement, nous les connaissons ! Elles s'adressent toutes aux mêmes personnes : les salariés, à qui l'on va demander de faire des efforts supplémentaires. On ne réfléchit pas, on ne regarde pas s'il y a d'autres solutions, on a d'ores et déjà décidé que l'on demanderait aux salariés des efforts supplémentaires. Or, monsieur le rapporteur, puisque nous avons rédigé ensemble un rapport sur l'emploi des seniors,

En tant que rapporteure générale, je soutiens la proposition de notre collègue René-Paul Savary. Tout

Le scrutin est clos.

de la branche vieillesse, nous donne l'occasion de revenir sur l'annonce par le Président de la République de l'allongement de la durée de travail et de son projet de réforme des retraites, au nom des générations futures. En 2021, le déficit de la branche vieillesse a reculé de 900 millions d'euros, malgré l'augmentation des dépenses, pour atteindre 4 milliards d'euros. Les prévisions les plus pessimistes prévoient un déficit de 7 milliards d'euros en 2025.

Le Gouvernement et la majorité sénatoriale parlent de la nécessité de s'attaquer à notre système de retraite en allongeant la durée de cotisation, ce qui va pénaliser les salariés de notre pays et en premier lieu les femmes, qui assument qui assument les congés maternité et subissent les inégalités salariales. Nous refusons ce recul social au nom d'un déficit de 1 % du budget de la sécurité sociale. Je mets aux voix

de programmer l'affectation de ressources publiques nouvelles destinées à soutenir la croissance des besoins de la branche autonomie. De nombreuses possibilités de financement existent : elles sont énumérées dans le rapport de Laurent Vachey en 2020 comme dans le rapport remis par la CNSA. L'un comme l'autre ont dessiné des pistes afin de programmer les ressources nouvelles nécessaires pour soutenir à long terme les politiques publiques en faveur de l'autonomie. Pour notre part, nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement

L'amélioration des hypothèses macroéconomiques se traduit par une augmentation des dépenses du FSV au profit des régimes de retraite, au titre de la prise en charge des cotisations.